de la mission d'information sur le thème : « Protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale écologique du XXI siècle. » Conformément à l'article 8 du règlement, les listes des candidats remises par les groupes politiques ont été publiées. Elles seront ratifiées s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle la suite

de 1,9 milliard d'euros, en cohérence avec l'actualisation du scénario macroéconomique ; d'autre part, traduire dans le tableau d'équilibre l'incidence des votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie

pour tenir compte de la révision à la hausse des hypothèses macroéconomiques du PLF et de plusieurs informations nouvelles. J'avais annoncé au cours de la discussion générale que le Gouvernement envisageait de modifier les hypothèses macroéconomiques. Conformément à l'article 16 de la loi organique du 17

les recettes fiscales sont majorées de 1 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros sur l'impôt sur les sociétés et 1,1 milliard d'euros sur la TVA, ces hausses étant partiellement compensées à hauteur de 600 millions d'euros par l'actualisation à la baisse d'autres taxes intérieures de consommation, ainsi que par l'actualisation du taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires. D'autre part, les recettes non fiscales sont majorées de 900 millions d'euros pour prendre en compte de nouvelles informations, à savoir la hausse des recettes relatives aux participations de l'État pour 600 millions d'euros et le remboursement du trop-perçu par Île-de-France Mobilités (IDFM), initialement prévu en 2021, pour 300 millions d'euros. ailleurs, les votes intervenus lors de l'examen de la première partie du texte au sein de votre assemblée ont eu pour conséquence de dégrader les recettes de 2,8 milliards d'euros. Les recettes fiscales brutes semblent minorées de 100 millions d'euros pour tirer la conséquence sur les recettes de la TVA de la création d'un taux réduit de 5,5 % appliqué à la margarine.

L'article d'équilibre retrace l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre, comme le dirait notre excellent collègue Vincent Delahaye, entre les recettes et les dépenses budgétaires. Le déficit budgétaire de l'État s'établissait, selon le projet de loi de finances initial, à un niveau de 143,4 143,4 milliards d'euros, financé par un emprunt de 260 milliards d'euros. Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, la prévision de déficit a été aggravée de 12 milliards d'euros supplémentaires pour atteindre 155,1 milliards d'euros. est due, notamment, à l'avalanche de nouvelles mesures annoncées depuis trois mois, autant de chèques en bois distribués à toutes les catégories de Français, à quelques mois de l'élection présidentielle. Pourtant, Emmanuel Macron ne déclarait-il pas en 2018, qu'« il n'y a pas d'argent magique » ? Certes, la crise a nécessité d'augmenter certaines dépenses pour répondre à l'urgence et relancer notre économie.

que 2021 marque la « sortie du quoi qu'il en coûte ». C'est le cas. Vous aviez même ajouté : « Le niveau de dépenses que nous connaissons aujourd'hui n'est pas soutenable dans le temps », ce que nous savons tous. Bruno Le Maire, au mois d'août 2021, avait lui aussi déclaré : « Le quoi qu'il en coûte, c'est fini !

N'ayant pas la possibilité technique ni même juridique d'établir un contre-budget, nous ne pouvons pas, en responsabilité, cautionner une telle dérive de dépenses, qui ne fait qu'accroître encore plus le déséquilibre budgétaire et aggraver notre endettement, à l'heure où les taux d'intérêt pourraient remonter.

Ce projet de loi de finances comporte finalement assez peu de mesures porteuses de recettes, à l'exclusion du bouclier fiscal introduit à l'Assemblée nationale en réaction à la hausse des prix de l'énergie. Le budget que vous nous proposez, monsieur le ministre,

que la situation sanitaire reste suffisamment maîtrisée pour que nous n'ayons pas collectivement à réactiver des dispositifs d'urgence particulièrement coûteux, mais particulièrement utiles ; tout le monde l'a reconnu et les a votés.

de vote sur l'article. Le constat est sans appel : la majorité sénatoriale a décidé de saboter l'examen de la seconde partie la réduisant à peau de chagrin. Nous venons d'examiner la première partie du budget. En refusant d'adopter l'article d'équilibre, nous ne pourrons pas débattre de la deuxième partie sur la répartition des crédits. Autrement dit, le Sénat n'examinera pas le budget dans son intégralité. Jusqu'à aujourd'hui, il me semblait impensable d'examiner les recettes d'un budget sans pouvoir débattre de ses dépenses. Cela me semble manquer d'audace et témoigner d'une incohérence déconcertante. vous n'avez cessé de dire que ce budget était incomplet. Or, aujourd'hui, il l'est effectivement. Par conséquent, je m'interroge. Que pensez-vous de la répartition des crédits ? Quelles économies feriez-vous ? Quelles seraient vos propositions d'ajustement ? En choisissant une telle stratégie, vous optez en réalité pour la facilité. Vous vous privez de modifications qui auraient pu être pertinentes. Vous nous privez de la possibilité d'ajuster les dépenses de ce budget. Vous privez tout simplement notre assemblée de pouvoir débattre en séance publique. de prise de position, vous ne ferez aucune proposition sur les dépenses sans parler de votre silence ahurissant lors de l'examen de la première partie

sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2022, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, chacun des groupes dispose de cinq minutes pour ces explications de vote, à raison d'un orateur par groupe. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

Il est difficile d'envisager un avenir serein dans ce paysage incertain. La situation ne permet pas encore d'entrevoir une quelconque sortie de crise. Si le Haut Conseil des finances publiques se dit lui-même incapable de rendre un avis sur ce budget, comment pourrions-nous le faire ? Nous avons suivi assidûment les prises de parole du chef de l'État et de son gouvernement. Nous nous sommes réjouis de l'intérêt accordé à la jeunesse, aux indépendants, à Marseille, à la police, mais nous avons aussi été surpris par ce plan d'investissement faramineux de 34 milliards d'euros, dont 3,5 milliards d'euros pour l'année 2022. Surtout, ces mesures ne sont pas toutes intégrées au budget ou l'ont été tardivement par voie d'amendements. Par exemple, le plan France 2030 est apparu par le biais d'un amendement qualifié comme « le plus cher de la V République ». Face à un texte qui manque de clarté et devant un budget à trous, nous ne pouvons pas nous prononcer sur ces mesures de façon juste et pleinement éclairée. Nous exigeons de la transparence. Nous ne pouvons pas jouer avec l'argent des Français, qui s'inquiètent de jour en jour de la diminution de leur pouvoir d'achat. La pauvreté ne cesse de gagner du terrain en France, malgré une reprise économique que je ne conteste pas. Nous n'aurions pas été contre plus de justice sociale, plus de justice fiscale et plus de justice écologique. Nous n'aurions pas été contre une meilleure attribution des crédits sur l'emploi, sur l'aide alimentaire et sur l'hôpital public. Soignants comme enseignants démissionnent faute de considération pour leur travail et d'augmentation de leur salaire. Quelles sont les véritables mesures pour pallier leur désespoir ? Nous souhaitons des solutions concrètes et pérennes sur la hausse des prix de l'énergie, sur l'urgence environnementale et sur le développement des énergies renouvelables. Nous ne voulons pas de réponses ponctuelles, prises dans l'urgence, à des problèmes qui risquent de perdurer.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce n'est un mystère pour personne : la majorité sénatoriale va rejeter la première partie de ce projet de loi de finances et empêcher ainsi l'examen du volet consacré aux dépenses. Nous partageons le constat que le Gouvernement ne respecte pas le Parlement, en introduisant des milliards d'euros de crédits par voie d'amendements après l'adoption de son projet à trous en Conseil des ministres. Le Haut Conseil des finances publiques l'a fermement dénoncé au mois

Ces derniers jours, j'ai entendu la droite s'élever contre l'absence d'économies réalisées dans le budget. Quel dommage dans ce cas de ne pas étudier la partie sur les dépenses ! Je suis sûr que vous n'auriez pas manqué d'idées pour réduire le déficit en diminuant certains crédits. Vous nous laissez sur notre faim Avec mes collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, nous regrettons un tel choix, qui prive notre assemblée d'une de ses missions essentielles : l'examen du budget dans son intégralité. Chers collègues du groupe Les Républicains, n'êtes-vous pas plutôt gênés par le fait que le Gouvernement présente un budget dont vous partagez en réalité les grandes orientations ? Bruno Le Maire l'a dit lui-même, la semaine dernière : « Certains candidats de la droite en ont rêvé, nous l'avons fait pendant ce quinquennat ! » Il a dit cela sérieusement ? Et, en effet, ce budget est de nouveau marqué par l'entêtement du Gouvernement à ménager les plus riches de nos concitoyens comme les grandes entreprises.

de solidarité sur la fortune (ISF) n'avait pas accru l'investissement productif dans notre pays. Au printemps dernier, Jean Pisany-Ferry et Olivier Blanchard plaidaient pour une rallonge de 60 milliards d'euros au plan de relance, dont une partie pour venir en aide aux ménages les plus modestes. Vous le voyez, monsieur le ministre, les alertes se succèdent, mais vous les ignorez encore et toujours. C'est sûr ! Vous persistez à mettre en oeuvre votre politique de l'offre « quoi qu'il en coûte ». Quoi qu'il en coûte sur le plan budgétaire, avec l'accroissement du déficit public Quoi qu'il en coûte sur le plan social, avec l'augmentation des inégalités, la baisse du pouvoir d'achat des Français les plus modestes, mais aussi la menace du retour de l'inflation et l'explosion des prix de l'énergie

et, pour les jeunes, des contrats d'engagement réduits aux acquêts. Sans compter que les grandes dépenses sacrifiées depuis 2017 correspondent pour l'essentiel aux ministères chargés de la solidarité et de la cohésion territoriale. Oui, il faut veiller à la compétitivité de notre pays ! Mais celle-ci ne peut pas se résumer à la fiscalité du capital, et votre politique reste déséquilibrée. Aujourd'hui, vous vous obstinez à la reprendre, comme si de rien n'était, alors que le moment est marqué par tant d'incertitude, et en faisant reposer tout le coût de la crise sur les Français. Nous pensons vraiment que c'est une erreur. Notre nation doit dégager les moyens pour financer ses investissements d'avenir, ses services publics et sa transition écologique.

La parole est à M. Didier Rambaud, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la majorité sénatoriale, qui vient de rejeter l'article d'équilibre, nous prive du débat sur la deuxième partie du projet

et de respecter la fonction première du Parlement : le débat.

chaque fois, vous ne pouvez pas vous résoudre à supprimer des dépenses spécifiques, mais, à chaque fois, vous refusez d'en assumer les conséquences. Vous nous l'avez encore démontré mercredi dernier au sujet de l'indemnité inflation.

Et vous nous proposez de revenir la semaine prochaine pour des débats improvisés sur vos priorités de campagne, sans assumer les conséquences de votre position, plutôt que de discuter du budget de l'État.

totalement étranger. Le suspense est insoutenable : nous allons enfin savoir si la majorité sénatoriale veut, ou non, adopter ce budget ... En l'occurrence, nous avons assisté à un double discours assez troublant. D'une part, on a entendu tout le mal que certains pensent du texte, qu'ils jugent insincère et incomplet. D'autre part, aucune mesure majeure du projet de loi de finances n'a été supprimée, et rien ne justifie finalement que l'on s'y oppose.

la filière et d'envoyer un message clair à tous les acteurs économiques de nos territoires : « faire filière ». Nous avons voté plusieurs mesures fiscales importantes pour renforcer la résilience de nos installations agricoles, notamment celles qui exercent sous la forme de coopératives. Pour nos agriculteurs, particulièrement pour nos viticulteurs, ces mesures sont autant de signaux positifs que nous leur envoyons après cette année marquée par le gel.

que j'ai eu l'honneur de rapporter avec notre collègue Jean-François Rapin. À cet égard, notre position était claire : puisque les crédits suivent l'évolution prévue par la loi de programmation, qu'ils sont en augmentation et en phase avec les immenses enjeux qui se présentent à notre pays, nous avons proposé de les adopter.

un soutien décisif à ces communes. Sur ce sujet d'importance pour nos collectivités et pour notre ruralité, comme sur tant d'autres, nous gagnerions à poursuivre les débats jusqu'à leur terme : les jeux politiciens n'aident en rien.

de tenir la politique. C'est à la politique, au sens que l'on donne à notre action, qu'il revient de tenir la technique. Oui, nous avons voulu sortir pour une fois du train-train budgétaire et affirmer un certain nombre de vérités ! Le vote auquel nous allons procéder aujourd'hui

Monsieur le ministre, le budget que vous défendez est indéfendable, car c'est un budget de campagne électorale, et de la campagne électorale la plus chère de la V République ! Eh

une véritable réforme des retraites. Voilà un Président de la République qui avait promis au pays une cure de jouvence et un monde nouveau. Or il utilise les plus vieilles ficelles de la classe politique depuis quarante ans : toujours plus de dépenses publiques ! Un problème

pour la justice dans notre pays, pour financer la solidarité et la transition écologique ! La parole est à M. Pascal Savoldelli,

d'un simulacre d'alternative, alors que vous avez toujours voté les projets de lois de finances de ce gouvernement. La majorité sénatoriale parle d'« insincérité politique ». C'est difficilement crédible quand, dans le même temps, elle imagine à la hâte un dispositif de soutien au pouvoir d'achat qui ne concerne plus que 6,1 millions de nos concitoyens, alors qu'un autre en concernait 36 millions

pas moins de 149, sans compter les passerelles de consensus établies avec la majorité sénatoriale. En témoigne l'effet d'annonce d'un plan d'investissement de 34 milliards d'euros sans aucune garantie démocratique. Le dogme libéral irrigue la moindre ligne budgétaire de ce projet de loi de finances. Pour cette seule première partie, vous nous présentez des avantages fiscaux pour la transmission d'entreprises, des avantages fiscaux pour la cession de titre ou d'entreprise, des avantages fiscaux pour les grands propriétaires agricoles- mais il n'y a rien pour les petits propriétaires agricoles

Il aura fallu moins d'une journée de débats pour aboutir à un texte finalement dérisoire par rapport à des désaccords supposés et revendiqués entre la droite et la droite et entre la droite et le Gouvernement ! Autant dire que notre institution a été prise dans un étau qui ne fait pas grandir la démocratie représentative ! Cette triste prestation ne manquera pas d'alimenter les constats de l'écrivain Bruno Le Maire, qui souhaite- et c'est grave limiter les compétences du Sénat en matière budgétaire à des observations et à une approbation finale, et non plus à une lecture complète ». Cela reviendrait à réduire le Sénat à un rôle de consultant, sans pouvoir de proposition, et d'observateur de la politique du Gouvernement.

Tous les niveaux de collectivités voient leur panier fiscal profondément modifié », sans que les objectifs ayant présidé aux réformes soient toujours atteints. Nous souhaitions supprimer le prélèvement forfaitaire unique abaissant substantiellement la fiscalité des dividendes, ou encore- c'était attendu ! -rétablir l'ISF, symbole de justice fiscale et sociale. Quelques jours après la fin de la COP26, ce budget reconduit des niches fiscales coûteuses et nocives, ignorant ainsi l'urgence de réduction de nos émissions de CO2.

Je vous le dis clairement : être en responsabilité, c'est savoir dire non ! Être sincère, c'est avoir déposé la question préalable ! Notre rejet est de gauche, et il est aussi responsable que sincère !

le groupe Union Centriste a abordé la discussion de ce projet de loi de finances pour 2022 avec l'intention d'en examiner les deux volets : les recettes, dans un premier temps de la discussion qui s'achève aujourd'hui, mais également les dépenses, lesquelles concentrent la moelle de ce projet de budget. Nous exerçons, en tant que parlementaires, un rôle central pour le consentement démocratique à l'impôt et symétriquement, pour ainsi dire, un rôle cardinal d'autorisation, de contrôle et, de manière certes plus limitée, de détermination des dépenses de l'État. Il nous apparaît difficile de dissocier ces deux missions, dès lors que l'objet premier des recettes que nous avons examinées depuis jeudi dernier réside dans le financement de la dépense dont nous aurions dû débattre à compter de ce soir. Par cohérence, nous aurions donc souhaité aller au bout de cet ultime marathon budgétaire de la mandature. Dernier du quinquennat, ce budget est aussi celui qui signe la sortie de la crise sanitaire et le parachèvement de la relance économique. Compte tenu de l'état de délabrement de nos finances publiques, état lié tantôt à la nécessaire réponse de l'État à l'épidémie de covid-19, tantôt, il faut bien le dire, à un certain laisser-aller budgétaire de type préélectoral, notre groupe avait entamé l'examen du budget avec le souci de défendre une ligne budgétaire vertueuse. Du côté fiscal, nous avons proposé, dans le sillage de ce qui avait été avancé par le précédent rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, mais avec cette fois-ci un effet immédiat, de transformer l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en impôt sur la fortune improductive, afin notamment de réintroduire dans l'assiette fiscale de l'IFI le patrimoine polluant dit « luxueux » et, ainsi, de respecter les engagements environnementaux pris lors des accords de Paris. La taxation des voitures, yachts et autres avions est un enjeu écologique avant d'être un enjeu financier, et les imperfections de l'IFI mériteraient d'être gommées. En fait de convergence entre efficacité fiscale et préoccupation environnementale, nous saluons la création, sur l'initiative de notre collègue Vincent Capo-Canellas, d'un suramortissement pour l'acquisition d'avions peu polluants. De même, nous nous réjouissons de l'adoption d'un mécanisme anti-abus renforcé de lutte contre les montages frauduleux d'arbitrage de dividendes, qui nous auraient fait perdre en vingt ans au moins 33 milliards d'euros de recettes fiscales. Cette proposition, formulée au sein de notre groupe par Nathalie Goulet, le fut aussi par d'autres, preuve de la capacité du Sénat à transcender les clivages de manière intelligente et sereine. Je tiens ici à insister sur la qualité et la pondération des débats que nous avons eus, dans une atmosphère toujours courtoise. Les avancées obtenues par le Sénat, au travers d'amendements émanant de toutes les travées de l'hémicycle, L'examen de la première partie de ce projet de loi de finances a permis à notre groupe de récolter une jolie moisson, avec plus du quart des amendements adoptés. Outre ceux sur l'IFI et la fraude à l'arbitrage de dividendes, nous nous félicitons des amendements, peu dispendieux, mais fort utiles, adoptés sur l'initiative des membres du groupe Union Centriste en faveur des services à la personne, des veuves d'anciens combattants, des agriculteurs, des doctorants, ou encore de la filière bois. J'ai ici à l'esprit les amendements de mes collègues Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin, Pierre Louault, Laurent Lafon ou encore Michel Canévet. Une autre satisfaction pour nous a été de voir adopter des mesures en faveur des collectivités territoriales et de leurs élus, au travers d'amendements déposés par des membres de notre groupe siégeant à la commission des finances, notamment Bernard Delcros, Hervé Maurey, Jean-Michel Arnaud, Vincent Delahaye, Jean-Marie Mizzon et moi-même, qui me félicite tout particulièrement de l'augmentation de la dotation élu local. Nos regrets quant à l'arrêt prématuré de la discussion sont d'autant plus grands que nous avions, du côté des dépenses, des propositions à faire. Malheureusement, le débat semble devoir se clore là. Dans ces conditions, malgré les améliorations évoquées, les membres du groupe Union Centriste, dans leur unanimité, ne prendront pas part au vote de la première partie. Ce n'est pas très grave ! La parole est

d'un côté, par ceux qui sont pour la dépense publique et l'impôt- Éric Bocquet a dit qu'il fallait actionner le levier fiscal

Monsieur le ministre, vous aviez

lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

En conséquence, mes chers collègues, en application de l'article 42 de la loi organique du 1 août 2001 relative aux lois de finances et de l'article 47 de

l'ensemble des rapporteurs spéciaux de la commission des finances pour leurs rapports budgétaires, qui restent des documents de travail pour nous tous comme pour l'extérieur.